La séance est ouverte. Le compte rendu intégral de la séance du jeudi 6 janvier 2022 a été publié sur le site internet du Sénat. Il n'y a pas d'observation ? ... Le procès-verbal est adopté. l'éducation et de la communication, de la proposition de loi relative à la circulation et au retour des biens culturels appartenant aux collections publiques, présentée par Mme Catherine Morin-Desailly,

sur le nez ! -est obligatoire dans l'hémicycle, y compris pour les orateurs s'exprimant à la tribune, conformément à la décision de la conférence des présidents réunie le 1 décembre dernier.

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, le Sénat a toujours joué un rôle moteur dans la réflexion sur les modalités d'une gestion plus éthique de nos collections publiques. C'est la chambre haute qui fut à l'initiative, grâce à notre ancien collègue, Nicolas About, de la loi relative à la restitution par la France de la dépouille mortelle de Saartjie Baartman,

C'est le Sénat encore qui fut à l'initiative, dans le cadre de cette seconde loi, de la création de la Commission scientifique nationale des collections, pour encadrer les déclassements de biens appartenant aux collections et pour définir une doctrine générale en matière de déclassement et de cession. Notre ancien collègue Philippe Richert, rapporteur de cette loi et rapporteur en 2021 du projet de loi relatif aux musées de France, jugeait cet outil indispensable pour faire progresser la réflexion sur la possibilité d'aliéner des biens appartenant aux collections sans compromettre le patrimoine de la Nation.

n'a nullement avancé en raison des préventions manifestées par le ministère de la culture et par une partie des conservateurs, qui, il faut bien le dire, ont été formés d'abord pour garder les La Commission scientifique nationale des collections a même fait les frais de la politique de rationalisation du nombre des commissions consultatives et a été supprimée, sur l'initiative du Gouvernement, par la loi d'accélération contre notre volonté. Cette décision me paraît d'autant plus regrettable que je suis convaincue, avec mes collègues, que les problèmes de fonctionnement de la commission auraient pu être corrigés facilement par voie réglementaire. ce qui explique que nous nous retrouvions aujourd'hui sans aucune doctrine pour répondre aux demandes de restitution pendantes, et sans aucun garde-fou pour contrôler les velléités de répondre positivement et hâtivement aux demandes, qu'elles soient ou non Le mouvement des demandes de restitution n'a pas été correctement anticipé malgré les alertes lancées par le législateur depuis dix ans. Notre pays est donc acculé à prendre dans l'urgence des décisions dictées uniquement par des considérations diplomatiques, en contradiction avec les objectifs mêmes qui sous-tendent le principe d'inaliénabilité des collections. Cette situation a conduit la commission de la culture à engager en 2020, sous mon égide, un travail approfondi sur les questions du retour des biens culturels vers leur pays d'origine, afin de dresser le bilan de l'action de la France et de formuler un certain nombre de recommandations. Max Brisson et Pierre Ouzoulias, dont je tiens

Le retour des biens culturels n'est pas une question facile, reconnaissons-le, tant elle met en présence des enjeux multiples et souvent contradictoires. Elle suppose de parvenir à concilier le droit de chacun à avoir accès, dans son pays, à son propre patrimoine et au patrimoine commun de l'humanité, sans obérer les capacités de nos propres musées à remplir leurs missions. Les demandes de restitution questionnent la légitimité de la conception universelle de nos musées. Elles ébranlent le principe d'inaliénabilité des collections, qui constitue, depuis des siècles, leur colonne vertébrale, en prévenant le risque qu'elles ne soient dilapidées par la seule volonté du prince. La recherche d'une solution solide et pérenne pour répondre aux demandes légitimes de restitution est pourtant nécessaire. Les débats autour de cette question s'intensifient ces dernières années, notamment dans

l'Allemagne vient de consacrer des moyens financiers importants pour faire la lumière sur la provenance d'une partie de ses collections. Elle a par ailleurs conclu, il y a quelques mois, un accord avec le Nigéria en vue de lui restituer des centaines de bronzes du Bénin, présents dans ses collections et pillés par l'armée britannique à la fin du XIX siècle. Quant à la Belgique, elle est en passe d'adopter une loi-cadre pour faciliter la restitution des objets de ses collections qui ont été acquis de manière illégitime. Pour autant, il n'y a pas de réponse unique. D'une part, chaque pays a son histoire coloniale propre, et, d'autre part, nous n'avons pas tous le même régime de protection de nos collections et la solution retenue par tel pays n'est pas forcément transposable dans tel autre. C'est pourquoi la France doit absolument engager un travail de fond dans ce domaine,

Quelle méthode doit présider à l'examen des demandes de restitution ? Telle est la question qui nous est posée et à laquelle il nous faut répondre. Il est clair que la manière dont ont été conduites les dernières restitutions n'a pas été satisfaisante. Premier constat, le Parlement a été dépossédé de son pouvoir, ... Absolument ! ... alors qu'il est pourtant le seul habilité à autoriser la sortie de biens culturels des collections. Le législateur a la compétence exclusive de faire exception au principe d'inaliénabilité des collections, qui est de valeur législative. Malgré ce principe, soit le Parlement a été sollicité pour entériner la restitution de biens culturels que le Président de la République ou le Gouvernement s'était déjà engagé à rendre- ce fut le cas pour le sabre revendiqué par le Sénégal et pour le trésor d'Abomey revendiqué par le Bénin -, soit il a été contourné, dès lors que l'on a remis aux pays concernés les biens qu'ils revendiquaient sous la forme d'un dépôt. Ce fut la méthode retenue par le Gouvernement pour restituer, à la veille de dates symboliques

Deuxième constat, l'instruction des demandes a été menée dans une grande opacité, donnant le sentiment que les considérations diplomatiques l'emportaient sur tout le reste. Le travail scientifique que les musées ont effectivement réalisé pour instruire les demandes de restitution n'a, hélas, jamais été rendu public. Troisième constat, les pays demandeurs- ils nous l'ont dit -ont été frustrés par le processus. Ils observent un manque de clarté de la procédure et un déficit de concertation dans l'instruction. Le risque, à terme, est que les restitutions ne se résument à des opérations sans suite et ne se traduisent pas, comme nous le souhaitons, par le lancement de coopérations dans le domaine culturel et patrimonial, dont toutes les parties pourraient pourtant bénéficier. Pour éviter ces dysfonctionnements, il faut disposer d'une véritable méthode permettant de traiter les demandes de restitution avec la plus grande rigueur et la plus grande transparence, au plus près de la vérité historique. C'est le seul moyen de préserver le principe d'inaliénabilité des collections et de garantir une cohérence et une permanence aux décisions que notre pays sera amené à prendre sur les demandes de restitution, malgré les alternances politiques La proposition de loi dont nous débattons vise à nous doter d'une telle méthode, qui se veut avant tout transparente, collégiale et scientifique. L'article 1 vise à créer un Conseil national de réflexion sur la circulation et le retour des biens culturels extra-européens. Cette instance doit permettre de combler les faiblesses de la procédure actuelle, que nous avons identifiées, et de compenser l'inertie du ministère de la culture sur les questions de restitution.

premièrement, rendre un avis sur les demandes de restitution, afin d'apporter aux pouvoirs publics un éclairage scientifique dans leur prise de décision ; deuxièmement, mener une réflexion prospective en matière de circulation et de retour des biens culturels troisièmement, formuler des recommandations sur la méthodologie et le calendrier des travaux consacrés à la recherche de provenance des biens culturels conservés dans les collections publiques. La commission de la culture juge en effet essentiel qu'un coup d'accélérateur soit donné à la recherche de provenance d'un certain nombre de pièces de nos collections. Ce travail commence tout juste dans les musées et il s'agit clairement d'un élément crucial pour répondre correctement aux demandes de retour et aux questionnements actuels sur la légitimité de nos collections. C'est en connaissant mieux et en faisant mieux connaître le parcours des pièces qui composent nos collections que nous pourrons restaurer leur image et leur conception universaliste. Nous pourrons également démontrer ainsi que l'essentiel des pièces originaires de pays tiers n'a pas été acquis de manière illégitime.

pour tenir compte des problèmes de fonctionnement rencontrés par la Commission scientifique nationale des collections, le champ de compétences du conseil porte clairement sur les demandes de restitution et sa composition se trouve réduite à douze membres, ce qui garantira son efficacité. Il s'agit, pour l'essentiel, de personnalités qualifiées, choisies pour leurs

du jeu ces deux ministères de tutelle, tout en les incitant à engager une véritable réflexion sur ces questions. La création d'une instance scientifique pérenne apparaît opportune pour apporter plus de transparence à la procédure, pour recentrer l'examen des demandes sur la vérité historique et pour garantir une plus grande permanence dans les décisions de la France,

D'une part, il s'agit d'un véritable outil de protection pour éviter que les seuls intérêts politiques et activistes prennent le pas sur les considérations culturelles, historiques et scientifiques. Il s'agit également d'une protection contre les pressions dont les autorités politiques- nous en faisons partie - pourraient faire l'objet. S'il est vrai que les membres du conseil ne seront sans doute pas toujours experts des biens qu'ils auront à examiner, ils auront tout loisir d'entendre des spécialistes avant de rendre leur avis, comme le font les commissions parlementaires. Ils auront également l'obligation d'entendre le personnel scientifique du pays demandeur, afin d'assurer la bonne prise en compte de ses positions et de garantir la construction d'un dialogue propice à la mise en place de coopérations globales dans le domaine culturel et scientifique. D'autre part, ce conseil pourra contribuer à la formation progressive d'une doctrine en matière de restitution, sur la base de ses avis, ainsi que dans le cadre de la mission de réflexion prospective qui lui est dévolue. Cette mission pourra être menée de manière autonome ou en s'appuyant sur les saisines des ministres ou des commissions parlementaires dont le conseil fera l'objet. C'est la raison pour laquelle la commission estime que que la création de cette instance n'est pas du tout incompatible avec la perspective d'une éventuelle loi-cadre sur le sujet, puisque le Président de la République a confié à M. Jean-Luc Martinez une mission en ce sens, il y a quelques semaines. Nous ne savons absolument pas à quel moment ce travail pourra aboutir. Il y a un an encore, le Gouvernement estimait qu'une loi-cadre n'était pas envisageable et qu'il serait extrêmement difficile d'établir une critériologie suffisamment précise et exhaustive pour convenir à la multiplicité des cas susceptibles de se présenter. Il craignait que l'adoption de critères ne fasse obstacle à des restitutions qui seraient pourtant souhaitables. C'est en tout cas ce qui figure dans l'étude d'impact du projet de loi relatif à la restitution On peut s'interroger sur ce brusque revirement, compte tenu de l'état d'avancement du travail sur la recherche de provenance. La commission estime qu'il serait regrettable d'attendre l'adoption de ladite loi-cadre pour renforcer la transparence de la procédure de restitution et sa méthode. Le conseil national peut faire progresser de manière collégiale cette nécessaire réflexion sur les critères de restitution, dès à présent. La meilleure méthode

Si la loi-cadre vient à être adoptée, le conseil national se révélera utile comme instance de contrôle, dans la mesure où le Parlement ne sera alors plus saisi des différentes restitutions. J'en viens à présent à l'article 2, dont l'objet est de faciliter la restitution de certains restes humains conservés dans les collections publiques. Cet article a été intégralement réécrit par la commission lors de l'élaboration de son texte, même si l'objectif reste strictement identique. Le besoin de faciliter la restitution la restitution de certains restes humains est réel. Plusieurs pièces conservées dans les collections publiques mériteraient d'être restituées. Divers cas ont été portés à notre connaissance pendant les auditions, comme celui d'un groupe d'Inuits emmenés en Europe en 1880 pour être exposés dans des spectacles, morts de la variole, puis enterrés, et dont les squelettes ont été exhumés cinq ans plus tard à des fins de recherches scientifiques. Notre

a été mis en place par le ministère de la culture et le ministère de l'enseignement supérieur, à la demande de la Commission scientifique nationale des collections, pour examiner les voies possibles de restitution des restes humains sans avoir à recourir au vote de

a produit deux rapports, en 2015 et en 2018, qui ont permis de dégager un accord autour d'un certain nombre de critères de restituabilité. Sur la base de ces critères et de ceux qui avaient guidé l'examen de la loi relative à la restitution des têtes maories, l'article 2 définit un cadre général fixant la procédure et les conditions de restitution des restes humains par l'administration qui en est propriétaire. Il s'agit d'une procédure en deux étapes. La première, qui est destinée à faire automatiquement sortir des collections un certain nombre de restes humains, dès lors qu'ils répondent à une série de critères, se traduit par une inscription provisoire sur un inventaire transmis aux États d'origine des restes. La seconde prévoit la restitution par l'administration des restes humains, lorsqu'elle est demandée, sous réserve que ce retour réponde à une série de conditions supplémentaires. L'adoption de cette disposition constituerait une réelle avancée pour permettre à notre pays de répondre plus rapidement aux demandes de restitution portant sur des restes humains et pour accélérer l'identification des cas sensibles présents dans les collections. Il serait d'ailleurs important que les pays d'origine soient associés aux différentes étapes L'article 2 offre donc à notre pays une méthode pour traiter de cette problématique délicate selon un processus fondé d'un point de vue scientifique, ainsi que dans le respect de la dignité humaine et des croyances des autres peuples. Il permet de régler un certain nombre de cas

Je crois savoir que le ministère de la culture préférait la rédaction initiale de cet article, qui visait à créer une procédure judiciaire permettant, au cas par cas, l'annulation de l'acquisition par les musées de certains restes humains, en vue de leur restitution, comme l'avait préconisé le groupe de travail

très clair quant aux fragilités juridiques de ce dispositif, susceptibles de le rendre inopérant. En tout état de cause, il aurait fallu qu'un décret d'application fixe les critères pour permettre au juge de prononcer l'annulation. Or le fait que le décret d'application relatif à la disposition similaire qui figure n'ait toujours pas été publié, plus de trois ans après l'adoption du texte, nous a inspiré quelques craintes. Enfin, compte tenu de l'encombrement des tribunaux, nous avons estimé qu'il n'y aurait pas grand intérêt à transférer cette charge au juge. Par ailleurs, le juge administratif peut toujours être saisi en cas de restitution litigieuse par l'administration, ou même en cas d'inaction de sa part. C'est pourquoi la commission estime que la rédaction de l'article 2, telle qu'elle vous est soumise, constitue la meilleure voie pour avancer en matière de restitution de restes humains, un enjeu essentiel pour manifester la volonté sincère de notre pays de progresser en matière de gestion plus éthique de nos collections. Tel est donc le contenu des deux articles qui composent cette proposition de loi, dont l'objectif essentiel est de doter notre pays d'une méthode pour traiter les questions de retour et de circulation des biens culturels vers les pays d'origine. Elle s'inscrit en cela dans la continuité des réflexions

Madame la présidente, madame la rapporteure- chère Catherine Morin-Desailly -, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, je vous prie, au préalable, de bien vouloir excuser ma collègue Roselyne Bachelot, ministre de la culture, qui ne peut être avec nous cette après-midi compte tenu du changement d'ordre du jour, puisqu'elle participe au lancement du volet culturel de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, à Bruxelles, en ce moment même. Comme vous le savez, un travail considérable a été engagé depuis plusieurs années par le ministère de la culture sur la restitution de biens culturels des collections publiques, en particulier des oeuvres d'art issues du continent africain et d'un contexte colonial. Le Président de la République s'était prononcé, à Ouagadougou, en faveur du renouvellement et de l'approfondissement de la coopération culturelle entre la France et les pays africains. Il avait souhaité notamment que « d'ici à cinq ans, les conditions soient réunies pour des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain en Afrique ». Une première étape historique a été franchie, à la fin de l'année dernière, au service de cette ambition, grâce à l'adoption de la loi du 24 décembre 2020 relative à la restitution de biens culturels à la République du Bénin et à la République du Sénégal. Pour la première fois dans son histoire, la France a décidé le retour dans leur terre d'origine de biens culturels d'une valeur patrimoniale et symbolique de première importance pour les pays intéressés. Fait remarquable, le principe de cette restitution au Bénin et au Sénégal a été soutenu par l'ensemble des parlementaires, tous bords confondus.,

En quelques années, quel chemin a été parcouru ! Rappelons que, en 2016, le Gouvernement avait opposé un refus à la demande qui lui avait été adressée par les Béninois. Cette évolution est due à l'immense travail collectif qui a été mené par le Gouvernement, par les musées et bien évidemment par les parlementaires. Je veux particulièrement saluer l'implication du Sénat, qui a largement contribué, par ses réflexions, à éclairer les débats. Nous pouvons être fiers de cette loi, qui a d'ailleurs eu un grand retentissement en Europe, en particulier en Allemagne, en Belgique ou aux Pays-Bas, pays concernés par des problématiques comparables. Depuis sa promulgation, nos engagements ont été tenus de bout en bout. oeuvres du trésor d'Abomey ont fait leur retour au Bénin, en novembre dernier, après une dernière exposition à la fin du mois d'octobre, au musée du quai Branly-Jacques Chirac, dans le cadre d'une très réussie semaine culturelle du Bénin. Une cérémonie de restitution a eu lieu au musée, présidée par le Président de la République, avant la signature par les ministres de la culture français et béninois du transfert de propriété officielle au Bénin, le 9 novembre dernier. Une exposition aura lieu au printemps prochain, au Bénin. Quant au sabre dit « d'El Hadj Oumar Tall », son dépôt à Dakar par le musée de l'Armée a pris fin en décembre dernier, pour se transformer en transfert de propriété.

De nombreux séminaires de recherche se sont tenus sur la question, et nous avons procédé au recrutement de plusieurs chercheurs de provenance. Dans le même temps, des partenariats entre les musées français et africains se sont noués.

La ministre de la culture s'est ainsi récemment entretenue avec son homologue de Madagascar à ce sujet. Pour traiter ces différentes demandes, notre méthode reste la même. Elle consiste à mettre nos musées au coeur de l'instruction des dossiers et à instaurer un dialogue étroit avec le pays demandeur, afin de parvenir à une analyse partagée de l'historique des pièces restituées. cet historique qui permet de déterminer l'éventuelle origine violente de l'entrée des oeuvres dans les collections publiques nationales, laquelle est susceptible de justifier leurs restitutions. Or seul le travail des musées est en mesure de l'établir, lorsque c'est possible.

Chaque cas est particulier et s'inscrit dans une histoire coloniale particulière, mais il nourrit une réflexion globale. De même, les échanges renforcés entre les pays européens concernés par des demandes de restitution

ainsi que l'a souhaité le Président de la République, la proposition au Parlement d'un dispositif-cadre, qui permettra de procéder plus facilement, en fonction de critères définis précisément, à de nouvelles restitutions d'objets culturels issus du contexte colonial africain. Pour nous aider à concevoir un tel dispositif, le Président de la République a confié à Jean-Luc Martinez, ancien président-directeur du Louvre et ambassadeur pour la coopération internationale dans le domaine du patrimoine, une mission visant à approfondir les consultations que la loi de 2020 a permis d'entamer.

Tout d'abord, les musées et leurs experts doivent être au coeur du dispositif d'instruction des demandes de restitution et, plus largement, des politiques sur la recherche de provenance.

L'histoire des pièces et de leur arrivée dans les musées doit être au coeur de toute instruction. Cette dernière ne peut être réalisée avec précipitation, car elle doit s'inscrire dans le temps long de la recherche. Les éléments de doctrine et de contexte que je viens de rappeler à cette tribune expliquent l'opposition réitérée du Gouvernement à la création d'une instance extérieure aux musées, qui serait chargée de se prononcer sur les projets de restitution. Certes, nous partageons avec les auteurs de cette proposition de loi l'objectif d'associer les scientifiques et les experts pour éviter tout fait du prince- nous l'avons démontré dans le traitement des dossiers béninois, sénégalais et ivoirien

Leur place dans les musées peut se justifier, notamment certains restes archéologiques ou objets constitués à partir de restes humains ainsi transformés, comme dans certaines collections anthropologiques. Sur ce point, on ne peut qu'être favorable à l'article 2, puisqu'il entend délimiter assez strictement le champ des restes humains restituables.

porter atteinte au principe de dignité de la personne. Troisièmement, ces restes doivent appartenir à des groupes humains encore existants, dont les cultures sont actives, et leur restitution ne peut avoir comme finalité

celui d'un âge maximal des restes humains, pour que ceux-ci soient restituables. Il nous semble nécessaire de considérer qu'au-delà d'une certaine ancienneté, par exemple cinq un reste humain ne peut plus être restitué, car le lien avec le peuple d'origine apparaît forcément distendu et plus difficilement rattachable à une population actuelle.

Dernier point, l'élaboration d'une liste intermédiaire de biens restituables fragilise le principe d'inaliénabilité en instaurant une nouvelle catégorie, en droit, dans les collections publiques. répertoriées « Musées nationaux récupération », ou MNR, issues de la récupération artistique après la Seconde Guerre mondiale, ne saurait lui être comparé. Ces biens figurent en effet sur une liste à part, parce qu'ils n'ont jamais intégré la domanialité publique, et cela du fait que, à l'origine il y a eu dépossession illégale de leur propriétaire privé. S'agissant d'objets faisant partie intégrante des collections publiques, l'établissement d'une telle liste crée une catégorie dont le statut en droit paraît un peu nébuleux : ils ne sont ni dans les collections publiques ni vraiment en dehors ; ils possèdent en quelque sorte un statut d'attente. nécessiterait en outre un travail colossal, dans lequel le Muséum national d'histoire naturelle (MNHN), qui est le principal concerné, tout comme les autres musées de France qui ont des collections d'anthropologie physique, n'aurait certainement pas les moyens de s'engager. Il conviendrait, sur ce point en particulier, de consulter le président du MNHN, ce qui à notre connaissance n'a pas été fait. Dans ce contexte, malgré une volonté partagée d'aboutir un jour à un texte permettant de régler ce sujet spécifique et de faciliter les restitutions quand elles sont justifiées, le Gouvernement ne soutiendra pas, à ce stade, la présente proposition de loi.

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, la restitution des biens culturels est un sujet complexe, qui mêle des intérêts et des acteurs divers et bien souvent opposés et qui suscite de nombreuses interrogations,

Cicéron plaidait déjà en faveur d'une protection du patrimoine et de la restitution des oeuvres d'art spoliées à la province de Sicile par Verrès, gouverneur romain accusé d'abus de pouvoir et de vol d'oeuvres d'art. la saisie d'oeuvres d'art est le premier facteur de circulation des biens culturels. En 1815, après la défaite de Napoléon, les puissances alliées ont exigé le retour de plusieurs oeuvres subtilisées dans le cadre des campagnes militaires menées De la même manière, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en Allemagne, plusieurs des biens amassés par les nazis sont visés par des demandes de restitution. Les études sur la provenance des oeuvres dans les collections allemandes permettent de rendre certains biens culturels à des États étrangers, mais aussi à des particuliers, aux héritiers ou ayants droit des nombreuses familles juives spoliées par le régime nazi. Si l'on creuse la notion d'objet culturel, on s'aperçoit qu'elle se définit au travers de l'instrument juridique mobilisé et de la matière considérée : sa valeur peut être archéologique, artistique, scientifique, technique, religieuse, laïque, historique ou encore symbolique. Le bien culturel est porteur de sens ; il est la mémoire et l'empreinte de la culture dont il est issu. Il compose le patrimoine culturel d'une société qui lui permet de forger son identité, sa mémoire collective. C'est ce patrimoine culturel que l'on souhaite transmettre aux générations futures. Les écueils juridiques sont nombreux et mettent en lumière la particularité et la complexité du sujet.

à la Nouvelle-Zélande de la tête d'un guerrier maori, qui se trouvait depuis la fin du XIXsiècle dans les collections du Muséum d'histoire naturelle de Rouen. la décision du conseil municipal de la ville, qui ordonnait la restitution de la tête maorie à la Nouvelle-Zélande, a été annulée, sur requête du ministère de la culture, par le tribunal administratif de Rouen, qui s'est fondé sur le principe d'inaliénabilité des collections publiques.

qui, au début du XIX siècle, a été emmenée à Londres afin d'y être exhibée pour ses particularités physiques. Elle passa quatre ans au Royaume-Uni

ce retour. La question plus globale du devenir des restes humains conservés dans les collections nationales est toutefois restée durablement De même, si les instruments juridiques européens sont nombreux, notre droit se révèle aujourd'hui impuissant à faire face aux demandes de manière systématique. Le texte que nous examinons a vocation à pallier ces manques. On ne peut que s'en féliciter, surtout quand on sait que, selon le rapport établi par M. Felwine Sarr et Mme Bénédicte Savoy en 2018, quelque 90 % du patrimoine africain seraient conservés hors du continent. À mes yeux, l'histoire coloniale reste à écrire, à exposer, à expliciter. Elle relève encore d'un impensé qui ressurgira tant qu'elle ne sera pas prise en compte et abordée aux niveaux institutionnel et politique.

On ne peut pas évacuer la question des restitutions, qui met au coeur du débat le patrimoine, la culture et l'histoire et qui insuffle une nouvelle dynamique d'échanges et de respect. D'ailleurs, l'histoire récente en matière de restitution d'oeuvres

ont pris un nouveau tournant et que la réflexion sur la spécificité et les racines du bien culturel semble acquérir une nouvelle place dans le droit des restitutions. À défaut de la reconnaissance morale, voire philosophique, d'un droit des peuples spoliés, nous nous dirigeons vers une reconnaissance de la particularité des biens culturels. L'objet culturel a des racines, et ce sont ces racines qui doivent être reconnues et qui doivent présider à la décision conduisant au retour du bien. S'accrocher aux principes en matière de prescription des demandes ou à l'idée que nos collections nationales sont inaliénables ne peut plus être notre seule matrice. Pour aller plus loin, il faut créer les conditions, grâce à ce texte, mais aussi à d'autres dispositions à venir, pour que, dans tous les lieux détenant des oeuvres, il y ait une réelle anticipation des demandes de restitution. il conviendra de trouver la meilleure manière de conserver une trace de l'oeuvre artistique qui aura rejoint son territoire d'origine, sous la forme de photographies exposées, voire de copies, afin que la valeur symbolique et universelle de l'oeuvre d'art puisse continuer à être partagée par le plus grand nombre. Je tiens à souligner l'immense et excellent travail de la rapporteure Catherine Morin-Desailly, ainsi de nos collègues Max Brisson et Pierre Ouzoulias, que j'ai eu grand plaisir à côtoyer. Le texte que nous examinons aujourd'hui ouvre

L'art ne connaît pas de frontière ; sa vocation est universelle. Les collections qui remplissent nos musées forment un patrimoine accessible à tous. L'art se nourrit des arts, et nombre d'oeuvres sont issues d'une influence multiple, irréductible à une culture ou à une civilisation. En révolutionnant l'approche occidentale de l'art, l'art africain a engendré l'art moderne. La France possède dans ses collections publiques près de 90 000 oeuvres d'art africain. Dans des sociétés dépourvues d'écriture, l'art faisait office de livre, support de la parole et vecteur de traditions et de croyances. Alors que d'innombrables oeuvres en bois ou en terre ont disparu, des milliers d'objets du quotidien sortis des malles de missionnaires, de médecins ou d'administrateurs ont bénéficié d'une conservation et d'une mise en valeur exceptionnelle au sein de nos collections. Nos musées sont des bibliothèques pour toute personne qui sait voir au-delà de la matière brute et lire l'histoire, la tradition ou la grandeur d'un peuple, qui est symbolisée au travers d'une sculpture de bois tendre et de kaolin. La puissance fascinante d'un masque fang du Gabon, fabriqué loin des regards, dans la solitude de la brousse, et exhibé lors des rites d'initiation, a autant contribué à écrire l'histoire culturelle de l'humanité qu'une danseuse de Degas ou un mobile de Calder.

Ce texte est l'aboutissement des travaux menés au Sénat en décembre 2020. Il vient combler les lacunes entourant les procédures actuelles de restitution. Face aux revendications croissantes de nombreux pays, notre groupe partage la volonté des auteurs du texte et de la commission de la culture de doter la France des outils juridiques appropriés.

Le Parlement n'est pas une simple chambre d'enregistrement des décisions du Gouvernement. Il convient de rappeler que la richesse des débats et l'indispensable confrontation des idées et des valeurs de chacun sont des éléments essentiels de notre démocratie. L'article 1 prévoit d'instaurer une instance scientifique chargée d'émettre un avis sur les demandes de restitution, en amont de la réponse politique. Le Sénat avait avancé cette idée lors de l'examen du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels à la République du Bénin et à la République du Sénégal. Le futur Conseil national de réflexion sur la circulation et le retour de biens culturels extra-européens comportera douze membres et aura la possibilité d'associer des scientifiques issus du pays demandeur, afin de contribuer à la réflexion. L'essentiel des oeuvres n'a pas vocation à être rendu à leur pays d'origine, mais un travail de fond sur la recherche de la provenance des oeuvres sera effectué au cours des prochaines années.

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, nous ne serions pas dans l'hémicycle ce soir sans le travail acharné de notre collègue Catherine Morin-Desailly. Je veux saluer la constance avec laquelle elle porte au Sénat la question de la circulation des biens culturels. Elle le fait sans jamais se départir d'une ligne directrice : donner à notre pays des règles claires et protectrices sur un sujet où la raison devrait toujours l'emporter sur la passion. Je souhaite également saluer Pierre Ouzoulias pour son travail et sa participation à l'élaboration d'un point de vue équilibré et constant. Ensemble, nous avons rédigé un rapport d'information à l'origine de la proposition de loi dont nous débattons aujourd'hui. Celle-ci s'inscrit dans le cadre d'un quinquennat qui fut marqué sur le sujet par une rupture politique majeure. Rappelons en effet que, à Ouagadougou, en 2017, le Président de la République affirmait : « Je veux que d'ici cinq ans- nous y sommes ! -les conditions soient réunies pour des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain en Afrique ». Dans le prolongement de ce discours, en novembre 2018, le rapport Savoy-Sarr recensait 46 000 oeuvres d'art provenant d'Afrique, susceptibles d'être rapatriées. inquiéter, semblait inexorablement lancé. Fort heureusement, le Président de la République s'est heurté à un obstacle de taille : le droit français. Bien sûr, sa volonté de restituer des oeuvres d'art n'est ni une nouveauté ni une singularité de ce quinquennat. Toutefois, la manière employée fut parfois pour le moins singulière, sinon déroutante, en particulier lorsque, pour répondre aux problèmes diplomatiques du moment, il a été procédé, sur ordre du chef de l'État, au transfert d'un bien sous couvert de prêt, plaçant la communauté des musées devant le fait accompli. C'est ainsi que le Gouvernement a renvoyé en catimini la couronne du dais de la reine Ranavalona III aux autorités malgaches. C'était au moment même où nous discutions, ici, du projet de loi de restitution des oeuvres au Bénin et au Sénégal. J'avais alors, tout en émettant des réserves sur ce projet de loi, appelé à établir une méthode pour aborder cette question avec recul et distance. Mme Roselyne Bachelot avait balayé fermement cette proposition. Certes, au Sénat, nous entendions et entendons toujours la demande des pays africains. Nous ne la contestions pas et ne la contestons toujours pas. Mais nous étions et nous demeurons profondément mal à l'aise d'observer le Gouvernement céder à une vision moralisatrice de notre histoire, tel que l'impose le rapport Savoy-Sarr, dont on sait combien il a faussé le débat. Nous aurions tellement préféré que le Gouvernement restât fidèle à l'héritage du président Jacques Chirac, lui qui avait chevillé au corps le dialogue des cultures. Oui, en lui étant fidèle, l'après-discours de Ouagadougou aurait pu être pour la France le moment de l'élaboration d'une véritable politique d'échanges et de circulation, qui aurait apporté une ligne de conduite constante sur un sujet ô combien important. Rien de tout cela ne s'est produit, bien au contraire ! En juin dernier, coup de théâtre : le Président de la République, prenant ministres et conseillers à rebrousse-poil de toutes les déclarations ministérielles antérieures, annonçait la nécessité d'une loi-cadre sur le sujet des restitutions ; Mme Roselyne Bachelot avait dit le contraire à cette tribune. Lorsque l'on parle de loi-cadre sur les restitutions, il faut d'abord rappeler que, pour nous, toute restitution est un cas à part. Voilà pourquoi le Sénat a toujours estimé que c'était au Parlement de se prononcer en dernier ressort sur chaque cas, mais que, pour cela, il devait être éclairé par un travail de recherche qui permette, pour chaque oeuvre, d'en connaître le parcours et, par l'intervention d'experts, le contexte ayant présidé à son dépôt et à sa conceptualisation artistique. La démarche présidentielle a donc enclenché un nouveau processus, bien tardif. L'ambassadeur thématique Jean-Luc Martinez a été désigné pour réfléchir au sujet. Malheureusement, au moment de son audition, nous n'avons pu connaître le contenu de sa lettre de mission. De même, l'exécutif, auditions après auditions,

nous avons été confortés dans ce que nous ressentions, à savoir combien est important le travail méthodique d'éclairage, de contextualisation, de recherche de provenance de chaque objet combien est important ce travail en coopération avec les scientifiques des pays demandeurs ; combien cela pourrait faire tomber les visions idéologiques visant à soumettre l'histoire de chaque oeuvre au prisme d'une vision globale empruntant les lunettes déformantes du présent pour la soumettre aux exigences présupposées de notre époque. Oui, chaque objet a une histoire propre, qui ne peut se réduire à une vision généraliste et être passée sans dégât au tamis de nos débats du XXI siècle. Ce travail minutieux, nous le devons au respect de la vérité historique. Or, justement, se doter d'une institution permettant d'élaborer un éclairage historique, historique, archéologique et muséologique, tel est l'objet de l'article 1 de la proposition de loi que j'ai l'honneur de porter avec Catherine Morin-Desailly et Pierre Ouzoulias.

Par cette proposition de loi, le Sénat quant à lui compte s'inscrire dans une position constante : la nécessité d'une analyse objective du contexte d'acquisition, fondée sur une méthode partagée. cela, le fait du prince continuera de sévir au service de la diplomatie, mais plus encore de la réécriture de notre histoire dans sa globalité, ... Ah ! ... ainsi que de l'histoire de chaque objet, soumis, malgré lui, à l'instrumentalisation politique de notre siècle.

madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, le 28 novembre 2017, devant les étudiants de l'université de Ouagadougou, le Président de la République prenait un engagement qui se voulait fort. Lors de ce discours, il reconnaissait qu'il était inacceptable que l'Afrique soit dépossédée d'une large partie de son patrimoine culturel et s'engageait à permettre, d'ici à 2022, « des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain en Afrique Voilà tout juste un an, nous examinions un projet de loi actant le retour du trésor de Béhanzin et le sabre avec fourreau dit « d'Oumar Tall », respectivement au Bénin et au Sénégal. Nous sommes encore loin d'un processus dynamique d'une diplomatie culturelle plus active avec le continent africain. En prenant en compte les demandes émises par tous les pays et connues à ce jour- Tchad, Mali, Éthiopie, Madagascar, etc. -, ce sont en effet plus de 13 000 biens qui devraient être examinés comme « candidats au retour » sur leur terre d'origine. Le texte de l'année dernière a été le seul et unique du quinquennat en provenance du Gouvernement sur ce sujet. Certes, le cadre législatif ne facilite pas les choses, puisque chaque restitution émanant des collections nationales doit faire l'objet d'un texte de loi spécifique.

que l'usage de ces lois d'exception « limite à l'extrême les cas de restitution » et qu'il conviendrait d'amorcer des démarches plus durables et globales avec les pays concernés. Il y a bien nécessité de sortir des lois d'exception et d'établir une coopération culturelle plus intense avec le continent africain. Cela passe par une forte évolution des mécanismes de restitution actuels, tributaires du fait du prince, souvent en dehors de toute considération scientifique ou patrimoniale. La présente proposition de loi va dans ce sens, ce que nous saluons. Ce texte prévoit la création d'un Conseil national de réflexion sur la circulation et le retour des biens culturels extra-européens. L'instance aura pour mission de donner son avis sur les demandes de restitution et sera composée d'experts de nombreuses sciences humaines et historiques chargés d'évaluer ces demandes. Nous espérons qu'il permettra d'objectiver les motivations des restitutions et d'en accélérer le processus- pressés de nous débarrasser de ce patrimoine, mais parce qu'il est temps de construire la coopération culturelle avec le continent africain sur des bases saines, affranchies autant que faire se peut des considérations purement diplomatiques ou politiques du moment. La proposition de loi procède d'une intention louable, la méthode est la bonne et elle pallie les manquements du Gouvernement.

et la nécessité d'un cadre stable de restitution. Oui, nous avons besoin d'un cadre stable pour ces restitutions. C'est le ciment indispensable d'une nouvelle approche avec le continent africain, une « nouvelle éthique relationnelle », comme le disent Felwine Sarr et Bénédicte Savoy. Le débat sur la dépossession de notre patrimoine culturel français est caduc. Il s'agit désormais d'instaurer un dialogue avec les pays d'origine de ces biens, afin qu'ils deviennent, comme nous l'avons été avant eux, les gardiens d'un patrimoine pour toute l'humanité. C'est cet idéal qu'il nous faut viser inlassablement, celui du dialogue entre chacune des cultures pour le bien de toutes et tous, celui du partage vu comme un enrichissement mutuel, et non une dépossession, celui de la justice et de la culture comme offrande faite au monde. C'est un combat de tous les instants, de toutes les politiques, fait de petits pas et de grandes avancées. La présente proposition de loi participe de ce mouvement. C'est pourquoi le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires votera en

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, « Est-ce là, où la religion ne permettait même pas aux hommes libres d'entrer pour prier, que tu as osé, toi, lancer les esclaves au pillage d'un sanctuaire ? Est-ce sur ces objets, dont le droit sacré te forçait à détourner même les yeux, que tu n'as pas hésité à porter les mains ? [ ...] Croyez-moi, juges, [ ...] si pendant ces dernières années nos alliés et les peuples étrangers ont subi nombre de malheurs et d'injustices, il n'en est pas qui soient et qui aient été plus pénibles pour des Grecs que ces pillages de sanctuaires et de villes ». Ainsi s'exprimait Cicéron lors du procès de Verrès, le gouverneur concussionnaire de la Sicile, qui avait pillé toutes ses oeuvres d'art. L'histoire des collections est souvent celle du vol, du dol, de la captation, du détournement ou de l'accumulation d'objets collectés sans grand souci de leurs origines et des conditions de leur réunion. Les temps ont changé, et il n'est plus possible de satisfaire la curiosité du public ou ses plaisirs esthétiques dans l'ignorance de leurs fonctions antérieures, des systèmes sociaux auxquels ils ont appartenu et des destins parfois tragiques qu'ils ont accompagnés. L'existence de ces objets et de ces oeuvres ne commence pas avec leur exhibition. Cette exigence éthique et scientifique de reconnaissance des circonstances des collectes est très loin d'être satisfaite pour une part majeure des oeuvres des collections nationales. Ce récolement général devrait être la première étape indispensable de toute démarche de restitution. C'est un travail de fond qui doit être réalisé de façon collégiale, par la mobilisation de plusieurs disciplines et en collaboration avec les scientifiques des pays d'origine de ces pièces. Disons-le sans ambages : au pire, il n'a pas commencé, au mieux, les moyens dérisoires qui lui sont consacrés éloignent d'autant son achèvement. Tant que cet inventaire ne sera pas suffisamment avancé, l'aliénation d'objets des collections nationales continuera d'obéir aux vicissitudes des petits arrangements entre États, aux sollicitations entre amis, aux traditions surannées des cadeaux diplomatiques, et il sera demandé au Parlement, tout en lui refusant le besoin d'en connaître, de voter sans renauder des lois de circonstance organisant dans l'urgence et la quasi-clandestinité leur dépossession. Il en fut ainsi des restitutions d'oeuvres au Bénin et au Sénégal. Le Sénat approuva leur principe, mais s'opposa, par une large majorité, à leurs modalités. Lors des auditions réalisées par notre commission pour l'examen de ce texte, il n'a toujours pas été possible d'appréhender les modalités d'instruction de ces demandes. Nous n'avons pas obtenu officiellement la copie des lettres adressées par les gouvernements du Bénin et du Sénégal, et il ne nous a pas été possible de déterminer pourquoi certaines oeuvres revendiquées par le Bénin ne lui ont pas été restituées. Ce retour des oeuvres béninoises aurait dû être le prétexte d'une collaboration culturelle ambitieuse entre nos deux pays. Il s'est plutôt apparenté à une froide opération notariale de transfert de propriété, qui a frustré les deux parties. Les restitutions devraient être l'un des éléments d'un échange culturel conçu comme un pont entre deux mondes qui regardent leur passé pour mieux construire leur avenir en commun. La forme législative appropriée de cette coopération pourrait être celle d'une convention internationale. Réduire la restitution à un article législatif constatant la radiation d'objets sur l'inventaire d'un musée est indigne de la valeur symbolique portée par les demandes. L'impéritie des services de l'État à engager le récolement des collections, l'absence de méthode pour l'instruction des demandes et le manque d'ambition politique et culturelle de la précédente loi de restitution ont conduit les signataires du présent texte à proposer la constitution d'un Conseil national de réflexion sur la circulation et le retour des biens culturels Constatant la nécessité de donner un nouvel élan à la politique de réparation des spoliations antisémites des oeuvres entre 1933 et 1945, le ministère de la culture s'est doté, en avril 2019, d'une nouvelle mission rattachée au secrétaire général du ministère. Sans confondre les deux offices, le Sénat considère que le conseil national proposé par ses soins a la même utilité pour insuffler, coordonner et rendre public les programmes d'échanges d'oeuvres. Vous nous expliquez, madame la secrétaire d'État, que les restitutions ne sont pas le fait du prince. Montrez-le

qui permettent une évolution nécessaire de la loi sur un sujet d'actualité récurrent. Le présent texte s'inscrit dans la droite ligne et la continuité des travaux menés de longue date par le Sénat sur ce sujet. Le groupe Union Centriste se mobilise sur la question depuis vingt ans. En effet, les deux premières lois de restitution de restes humains appartenant à des collections publiques françaises ont été adoptées sur l'initiative de Nicolas About et Catherine Morin-Desailly. Il s'agit de la loi du 6 mars 2002 relative à la restitution par la France de la dépouille mortelle de Saartjie Baartman à l'Afrique du Sud et de la loi du 18 mai 2010 visant à autoriser la restitution par la France des têtes maories à la Nouvelle-Zélande Dès 2007, Catherine Morin-Desailly a été mobilisée sur la question du retour des biens culturels. À cette date, alors qu'elle était adjointe à la culture du maire centriste de Rouen Pierre Albertini, elle avait fait adopter à l'unanimité pour restituer à la Nouvelle-Zélande la tête maorie appartenant au musée de la ville. Mais le ministère de la culture de l'époque avait contesté la délibération votée devant la juridiction administrative. Outre le texte législatif ponctuel qu'il aura donc fallu pour permettre ce retour, dès cette époque était apparue la nécessité d'établir une procédure et des critères objectifs pour traiter des réclamations étrangères de biens appartenant à des collections publiques. Faute de quoi, en dépit de leur protection par le principe d'inaliénabilité, les collections encourent un risque majeur d'arbitraire. Sans critère scientifique objectif, le fait du prince prévaut, ce qui revient à faire dépendre le sort des collections de l'aléa diplomatique. La loi de restitution des têtes maories avait mis en place une instance scientifique : la Commission scientifique nationale des collections (CSNC). Celle-ci était chargée de contrôler les déclassements et les cessions de biens appartenant aux collections publiques, ainsi que de définir une doctrine générale sur ces questions. La CSNC n'a toutefois pas joué son rôle, puisqu'elle s'est déclarée incompétente pour juger des demandes de restitution. Elle a été supprimée, sur l'initiative du Gouvernement, par la loi du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique. Le problème reste donc aujourd'hui entier. Mais il se pose avec plus de force que jamais, puisque les demandes de restitutions n'ont cessé de se multiplier au cours des dernières années. C'est bien ce qui a conduit le Président de la République à s'emparer du sujet lors du discours de Ouagadougou, le 28 novembre 2017, et à commander le rapport Sarr-Savoy. Cette actualité a accouché d'une troisième loi de restitution, la loi du 24 décembre 2020 relative à la restitution de biens culturels à la République du Bénin et à la République du Sénégal, qui concernait pour la première fois des oeuvres et objets d'art, non des restes humains. Le Sénat avait alors adopté un amendement visant à créer un conseil national chargé de réfléchir aux questions de circulation et de retour d'oeuvres d'art extra-occidentales. Cette création s'est opposée à un veto catégorique de la part du Gouvernement et de sa majorité. La CMP n'a pu aboutir en raison de cette mesure. Le 16 décembre 2020, en adoptant les conclusions de sa mission d'information sur la restitution des biens culturels appartenant aux collections publiques, le Sénat a formulé quinze propositions, qui constituent une doctrine unique en la matière. La présente proposition de loi concrétise les deux propositions faites par la mission d'information relevant du domaine législatif la création du Conseil national de réflexion sur la circulation et le retour des biens culturels extra-européens ; d'autre part, l'extension de la procédure judiciaire prévue à l'article L. 124-1 du code du patrimoine pour faciliter la restitution de certains restes humains appartenant aux collections publiques. La première de ces propositions, la plus importante, tire les leçons de l'échec de la CSNC, en donnant clairement compétence à l'institution créée de se prononcer sur les demandes de restitution et en resserrant sa composition autour de douze membres, au lieu d'un collège pléthorique. C'est le seul garde-fou possible pour éviter que les collections ne se transforment en « étagères à », dans lesquelles l'exécutif n'aurait qu'à piocher au gré de ses intérêts diplomatiques. Pour ce faire, le texte pérennise autant que possible le principe de l'inaliénabilité des oeuvres. Le patrimoine et l'histoire qui lui est associée ne doivent pas devenir des instruments politiques ou des variables d'ajustement dans les relations diplomatiques. Il s'agit, plus globalement, de réduire au maximum le risque d'arbitraire pesant sur les procédures de restitution. L'ambition de ce texte est de proposer un cadre précisant clairement les critères de restitution des oeuvres. Ceux-ci devront être déterminés de façon objective et scientifiquement établis. Nous nous réjouissons de voir que, au travers de cette proposition de loi, c'est l'humain qui prime. Nous affirmons nos valeurs. Les biens artistiques et culturels ne sont pas des biens comme les autres. Ils doivent respecter la dignité humaine et favoriser la transmission des valeurs entre générations.

affirme la « spécificité des biens et services culturels qui, parce qu'ils sont porteurs d'identité, de valeurs et de sens, ne doivent pas être considérés comme des marchandises ou des biens de consommation comme les autres ». Dans ces conditions, selon une conception identitaire, on peut comprendre la nécessité du retour d'un bien vers celui à qui il fait sens, tout comme on peut accepter la valorisation des biens culturels dans une perspective universaliste, car la culture s'épanouit au contact des autres. Bien entendu, au regard de notre histoire, en particulier de celle qui nous lie au continent africain, il est clair que ces deux approches peuvent se heurter. Aussi, la proposition de loi a le grand mérite de mettre en place un cadre rigoureux de nature à traiter, dans la transparence et sans arrière-pensées, les demandes de retour de biens culturels dans leurs pays d'origine. pays d'origine. Le RDSE est tout à fait favorable à son adoption. Madame la secrétaire d'État, ce débat peut-il ouvrir la voie à la loi-cadre voulue par le Président de la République ? La réflexion, en effet, ne sera pas épuisée aujourd'hui ... Au fond, quelle est la finalité du retour d'un bien culturel dans son pays d'origine ? S'agit-il pour le donateur de l'utiliser comme un levier de- « puissance douce », en français ? La multiplication des conventions de dépôt engagées par le Gouvernement participe sans doute au dialogue politique avec les pays d'Afrique. lorsque l'on sait qu'une grande majorité de biens culturels ont été acquis dans des conditions inacceptables, s'agit-il de faire acte de repentance ? On peut accéder à ce besoin moral de réparer, mais doit-on pour autant qualifier sans nuance les musées européens de « musées des autres », comme le fait le polémique rapport dit « Savoy-Sarr » ? À cet égard, dans le texte qui nous occupe ce soir, le choix du mot « retour », plutôt que celui de « restitution », va dans le sens d'un apaisement nécessaire autour de cette question sous-jacente des spoliations. Le retour fait référence à l'histoire et à la géographie, sans se focaliser sur les conditions d'acquisition. Pour le législateur, la meilleure façon d'éviter ces écueils est de mieux encadrer la politique de retour des biens culturels, en donnant avant tout un rôle accru aux experts, comme nous le faisons dans le présent texte. Pour autant, à terme, une réflexion plus vaste sera nécessaire. Comme l'a rappelé notre collègue Bernard Fialaire lors de l'examen de la loi relative à la restitution de biens culturels à la République du Bénin et à la République du Sénégal, le « retour » d'un bien culturel doit relever avant tout d'une réflexion culturelle. Le principe d'inaliénabilité, qui protège les collections publiques, apparaît bloquant, alors que, en réalité, il n'est pas absolu. En effet, ce n'est pas la nature d'un bien qui fait obstacle à l'aliénation ; c'est son affectation au domaine public. La procédure de déclassement le confirme. Dans une future loi-cadre, on attend un dépassement de ces notions. En réponse à des demandes de pays qui auraient un attachement historique ou identitaire à des biens culturels, il faut mettre en avant la notion de don, qui intègre l'idée de la propriété inaliénable du bien culturel au niveau de son essence, et non de sa matérialité. Ce droit doit en effet se construire à partir de la dimension culturelle d'un bien, pour dépasser son titre de propriété. Très bien ! Certains biens ont d'ailleurs acquis une vocation culturelle en sortant de leurs frontières, en se confrontant avec d'autres cultures. Cela relativise l'endroit où ils se trouvent. Une oeuvre a une vocation universelle et elle appartient au patrimoine universel de l'humanité, qui pourrait en être le nu-propriétaire. L'usufruit, quant à lui, trouverait sa place en fonction de son intérêt culturel, soit dans un musée à vocation universelle de dialogue interculturel, soit dans son pays d'origine si sa présence est nécessaire à l'approfondissement de l'identité de ce pays. La circulation des biens serait ainsi facilitée, sous réserve de l'amélioration des politiques muséales ou de conservation des pays d'accueil des biens culturels. Le corapporteur spécial de l'aide publique au développement que je suis ne serait pas opposé à un véritable renforcement des moyens de la coopération en matière d'ingénierie culturelle. En attendant, mes chers collègues, dans le sillage de Bernard Fialaire, le RDSE approuvera ce texte visant à un dépassement des frontières, à un patrimoine culturel partagé et à une meilleure concorde entre les peuples.

à de trop nombreuses reprises depuis cinq ans, le pouvoir exécutif a fait peu de cas de la représentation nationale et de la souveraineté du Parlement. En matière de patrimoine aussi, le Gouvernement s'est montré peu soucieux du rôle des parlementaires dans la préservation et la sauvegarde de nos collections nationales. Oubliant qu'elles ne lui appartiennent aucunement, le chef de l'État a pris la mystérieuse habitude d'agir seul et discrètement pour traiter les demandes de restitution, métamorphosant le Parlement en chambre d'enregistrement. S'il est louable que la France se saisisse de la question de la circulation des biens culturels, les méthodes retenues par l'exécutif semblent plus que contestables. Outre le mépris affiché envers les assemblées, le pouvoir exécutif fait fi de l'expertise scientifique et de la voix des acteurs de la culture. Or on ne peut mesurer la pertinence et l'opportunité de telles démarches sur les seuls critères politiques, diplomatiques et- pourquoi pas ? -médiatiques. Fût-il éclairé, un Président de la République ne saurait être un monarque absolu. D'ailleurs, dans le royaume de France, même sous Louis XIV, les prérogatives royales étaient encadrées. À plusieurs occasions et en l'espace d'une seule année, les parlementaires ont été placés devant le fait accompli : entre novembre 2019 et novembre 2020, trois restitutions à des pays étrangers ont été effectuées. Ce sont autant d'humiliations pour le Parlement, qui détient pourtant des prérogatives exclusives pour autoriser la sortie définitive de ces biens. Nonobstant l'intégrité de nos collections, c'est donc aussi le principe de séparation des pouvoirs lui-même qui est ainsi bousculé. Lors de son déplacement à Ouagadougou, en novembre 2017, le Président de la République expliquait vouloir poser les jalons d'une nouvelle politique patrimoniale avec l'Afrique. Dont acte Mais encore faut-il ne pas tomber dans le piège du fait du prince, car ce n'est pas à un élu, quel qu'il soit, de déterminer l'avenir de nos collections publiques. Le patrimoine n'est pas politique et son sort ne doit pas fluctuer au gré des alternances et de l'air du temps. Ce texte aspire ainsi à éclairer scientifiquement et sur le temps long la gestion de nos biens culturels. La teneur et la portée symbolique de ces questions nous obligent à ne pas les traiter dans la précipitation. Elles exigent un travail long et collectif de coopération avec les pays demandeurs. Chaque requête, d'où qu'elle vienne et quelle que soit sa nature, doit être examinée au cas par cas, car le seul contexte colonial ne peut suffire- tant s'en faut -à fonder la légitimité du retour d'un bien culturel, auquel cas l'ensemble de ces démarches s'assimileraient à des actes de repentance ou de contrition. ... Si l'histoire et les conflits de mémoire sont au coeur de ce débat, leur dimension passionnelle ne doit pas nous faire oublier un principe essentiel, multiséculaire, qui a été rappelé précédemment : l'inaliénabilité de nos collections publiques. C'est ce principe qui, depuis l'édit de Moulins de 1566,

Inscrire dans la loi cette instance de réflexion contribuerait à consacrer ce principe et à s'assurer que la circulation des oeuvres ne soit pas laissée à la seule discrétion d'un chef d'État dirigiste et peu scrupuleux du droit, malgré des arrière-pensées peut-être louables.

Une instance comparable existe d'ailleurs d'ores et déjà pour les questions relatives au patrimoine architectural. Depuis 2016, la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture est obligatoirement consultée dans le cadre de projets d'aliénation d'immeubles protégés au titre des monuments historiques appartenant à l'État. Cette consultation ne fonctionne pas forcément bien, Outre ce conseil de réflexion, le cas particulier de la restitution des restes humains, cher à Catherine Morin-Desailly, n'est pas à négliger. Ce ne sont évidemment pas des biens culturels comme les autres : c'est pourquoi il appartient au législateur d'aménager et de faciliter les procédures les concernant. C'est à cette fin que le Parlement doit consentir, dans le cas précis des restes humains et sur la base de critères stricts, à ne pas être systématiquement consulté. Vous l'aurez compris, madame la secrétaire d'État, cette proposition de loi a vocation à rappeler que nos choix en matière de circulation des biens culturels dépassent le champ diplomatique et les intérêts transitoires susceptibles de motiver la sortie d'une oeuvre de nos collections publiques. Aucune revendication mémorielle, nulle doléance communautaire ne doit déterminer, même partiellement, le sort de nos biens patrimoniaux. Le Parlement se devra toujours d'y veiller. je vous remercie

le bien de première importance que revendiquait le Bénin est la statue du dieu Gou, qui est restée au Louvre. Vous nous avez expliqué,

doit étayer la décision politique dans le cadre d'un débat public. L'origine des oeuvres, leur conceptualisation artistique, leur parcours doivent être connus.

Nous en sommes venus au temps où l'humanité ne peut plus vivre avec, dans sa cave, le cadavre d'un peuple assassiné. » Je le paraphraserai pour ma part ainsi : « Nous en sommes venus au temps où nos musées ne peuvent plus conserver dans leurs placards les crânes d'Arméniennes assassinées lors du génocide de 1915. » La parole est

Merci demande du groupe Les Républicains, de la proposition de loi visant à limiter l'engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée, présentée par M. Jean-Noël Cardoux et plusieurs de ses collègues

Ce phénomène n'est pas nouveau, mais il s'est accéléré considérablement depuis la loi de février 2005, laquelle- on se demande pourquoi ! -a permis aux propriétaires d'enclos attenant à une maison d'habitation de chasser le gibier à poil toute l'année, sans plan de gestion et sans contribution aux dégâts Avant 2005, il s'agissait d'un phénomène peu développé, motivé avant tout par une volonté de protection contre les intrusions ; après 2005, année de rupture, les enclos se sont multipliés, essentiellement pour pouvoir bénéficier des mesures dérogatoires, avec bien souvent des tableaux de chasse excessifs. Depuis deux ans, un tapage médiatique peu opportun a incité de nombreux propriétaires, craignant une interdiction, à se clore à titre préventif.

Voilà pourquoi la date de février 2005 a été choisie, en accord avec la Fédération nationale des chasseurs, qui soutient ce texte- je l'en remercie -, comme point de départ de la suppression des grillages existants, posés, pour la plupart, par opportunité cynégétique. Il faut néanmoins espérer que les territoires non concernés par cette date et ne pouvant plus bénéficier de dérogation engagent un désengrillagement volontaire, grâce à la mise en place, souhaitable, de mesures incitatives, en dehors des obligations réelles environnementales (ORE) : application stricte du plan de gestion forestière (PSG), bénéfice de l'écocontribution pour l'implantation de haies, exonération de taxe foncière.

doit toutefois permettre une prise de conscience, ainsi qu'une évolution rapide et irréversible. Il provoque des réactions opposées, certains jugeant qu'il va trop loin et d'autres pas assez ; j'en déduis qu'il s'agit d'un texte d'équilibre, raisonnable, posant des perspectives d'évolution. Au contraire des propositions de loi présentées à l'Assemblée nationale, il s'agit non pas d'interdire, mais d'équilibrer. néanmoins un virage fondamental, car, tout d'abord, elle respecte le code de l'environnement et la libre circulation des espèces dans les milieux naturels.

elle interdit en tout lieu l'engrillagement non franchissable par les animaux à partir de la publication de la loi. elle supprime les dérogations aux conditions de pratique de la chasse, quel qu'en soit le territoire. Enfin, elle offre une période de transition suffisante de

Ce texte prévoit une sanction, une contravention de cinquième classe, pour les pénétrations non autorisées dans les propriétés privées, qui est une contrepartie

de loi permet aussi aux gardes de l'Office français de la biodiversité (OFB) de pénétrer dans les territoires clos sans commission rogatoire, sauf dans les habitations.

de l'environnement, mais n'est pas sanctionnée, à défaut de décret d'application. En revanche, les schémas départementaux de gestion cynégétique permettent l'agrainage linéaire dissuasif à certaines périodes de l'année, pour une légitime protection des cultures ; nos amis agriculteurs le savent bien. La simple énumération de ces mesures montre le travail en profondeur effectué par tous ceux qui ont participé à l'élaboration de cette proposition de loi. Je remercie tout particulièrement Sophie Primas, la présidente de la commission des affaires économiques, Laurent Somon, notre rapporteur qui a eu un rôle moteur pour proposer des ajustements opportuns,

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, Jean-Noël Cardoux vient de vous présenter les raisons qui l'ont conduit à déposer cette proposition de loi et les principales dispositions Je voudrais tout d'abord le remercier, car c'est fort de sa très grande connaissance de la chasse, des milieux naturels et des espèces sauvages que nous pouvons examiner ce soir ce texte complet, équilibré et courageux, pour lutter contre l'emprisonnement de la nature, tout en assurant la protection de la propriété privée. Il s'agit aussi de s'opposer à l'artificialisation des milieux naturels et de défendre une chasse durable, éthique, exigeante et respectueuse des équilibres biologiques.

En tant que rapporteur pour la commission des affaires économiques, je voudrais insister sur deux aspects : l'esprit dans lequel nous avons travaillé et les compléments que nous avons apportés au texte, avec l'accord de son auteur. Sur ce texte, la commission a travaillé avec le souci du rassemblement, afin de faciliter sa future adoption à l'Assemblée nationale. Il m'a semblé qu'il ne fallait pas aborder la proposition de loi de manière partisane ou conflictuelle entre chasseurs et non-chasseurs, propriétaires et promeneurs, mais essayer de forger le consensus le plus large possible sur un sujet qui doit tous nous rassembler, même si certains voudraient aller plus ou moins loin sur tel ou tel point, j'en ai bien conscience. J'ai donc auditionné le maximum de parties prenantes. J'ai été frappé à la fois par les attentes très fortes de citoyens qui militent, parfois depuis trente ans, contre ce phénomène et par la maturité du débat et des solutions prêtes à être adoptées, Stevens et Michel Reffay, diligenté par le Gouvernement en 2019, a contribué à faire émerger. Cela explique que, en dehors de Jean-Noël Cardoux, trois collègues députés se soient également saisis du sujet : Guillaume Peltier, Bastien Lachaud et François Cormier-Bouligeon. Venant d'horizons politiques très différents, ils ont chacun, avec leur expérience de terrain, formulé des propositions et fait avancer la question. Je les ai rencontrés, car j'avais à coeur de les écouter, de tenir compte de leur travail et, autant que possible, de rapprocher le texte du Sénat des attentes d'ores et déjà exprimées à l'Assemblée nationale, car il nous faudra, dès que possible, aboutir à un texte commun. Dans le même esprit, madame la secrétaire d'État, j'ai travaillé avec vos services. J'ai pu prendre en compte leurs difficultés et leurs besoins pour assurer le contrôle et l'application de la loi, et ils m'ont apporté leur expertise. Je tiens à les en remercier. Ces travaux ont, en outre, été partagés avec des collègues d'autres groupes politiques, afin que nous puissions nous forger une opinion partagée. Cela s'est traduit en commission par le dépôt d'un certain nombre d'amendements identiques cela se traduira également, ce soir, par de nombreux avis favorables sur des amendements venus des différents bords de notre assemblée. Finalement, le texte qui vous est présenté ce soir a été largement adopté par la commission, traduisant la volonté d'avancer ensemble, malgré nos différences, vers une solution attendue pour mettre fin à l'engrillagement des milieux naturels. Forte de ce travail en partenariat que je viens d'expliquer, la commission a adopté plusieurs modifications au texte initial. Celles-ci résultent toutes d'observations et de demandes que nous avons recueillies lors des auditions et s'articulent autour de deux objectifs : mieux définir les caractéristiques des clôtures autorisées autorisées ; mieux assurer l'application de la loi, donc la lutte contre l'artificialisation des milieux naturels. Concernant tout d'abord les caractéristiques des clôtures, en se fondant sur des exemples concrets, la commission a été attentive à ce que celles-ci assurent le passage de la faune au sol et ne puissent ni blesser ni devenir des pièges pour les animaux. La commission a également précisé les exceptions pour lesquelles des clôtures hermétiques à la faune seront autorisées. Il s'agira des clôtures agricoles, sylvicoles et d'intérêt public. Concernant les clôtures sylvicoles, elles seront autorisées pour protéger la régénération de la forêt, mais pas dans le cas d'un massif sous plan simple de gestion, ce qui aurait été un dévoiement. Il semble, d'ailleurs, que beaucoup de zones actuellement engrillagées n'en respectent pas les prescriptions. S'agissant des clôtures d'intérêt public, il s'agit bien entendu d'assurer la sécurité des routes, des voies ferrées et des grandes infrastructures. On pourrait s'étonner que le législateur descende dans tous ces détails, mais l'élaboration d'une norme nationale résulte d'une large demande et apparaît aujourd'hui comme une nécessité pour aider les maires dans l'application des plans locaux d'urbanisme (PLU) ou les régions dans celle de leurs schémas d'aménagement. La commission s'est ensuite attachée à faciliter l'application de ces nouvelles dispositions. Elle a réduit de dix ans à sept ans le délai de mise en conformité, estimant que, si le premier était trop long, il ne fallait négliger ni les délais d'application de la loi ni les conséquences matérielles et pécuniaires de la remise en cause de droits légalement acquis ou d'exploitations commerciales. La commission a également souhaité favoriser l'effacement des clôtures antérieures à 2005, en permettant que l'écocontribution puisse être mobilisée pour les remplacer par des haies. Il était ensuite nécessaire de prévoir des sanctions en cas de refus d'appliquer ces nouvelles normes. La commission a estimé que l'engrillagement de la nature était assimilable à une atteinte au patrimoine naturel, aux milieux comme aux espèces, et qu'il devait être sanctionné comme tel dans le code de l'environnement. C'est pourquoi elle a retenu la possibilité de prononcer une peine maximale de trois ans de prison et de 150 000 euros d'amende. Cette peine apparaît proportionnée aux enjeux qui s'attachent à la clôture de grands territoires, laquelle n'est pas toujours motivée par la chasse. Dans les cas où cette dernière en est le mobile, l'engrillagement des espaces naturels pourra entraîner la suspension du permis de chasser du titulaire du droit de chasser. Par ailleurs, comme des enclos subsisteront pendant le temps de mise en conformité, ou, plus durablement, parce qu'ils sont antérieurs à 2005, la commission a voulu combler un vide en permettant aux agents de l'OFB de les contrôler sans se voir opposer la protection du domicile. Je vous proposerai tout à l'heure un amendement visant à étendre cette possibilité aux agents assermentés des fédérations. L'objectif est que, là où s'exerce la chasse, la police de la chasse puisse opérer sans entrave. En outre, il a paru nécessaire de compléter ces dispositions contre l'artificialisation des milieux et de la chasse, dont les enclos sont les archétypes, par une sanction en cas d'infraction aux règles d'agrainage et d'affouragement. Celle-ci pourra entraîner la suspension du permis de chasser du titulaire du droit de chasser. Enfin, la commission a souhaité accueillir favorablement la volonté des fédérations de chasseurs de s'impliquer plus fortement dans la police de la chasse, compte tenu des moyens limités de l'Office français de la biodiversité et afin de démultiplier ses efforts sur le terrain. Dans cet esprit, les compétences des agents assermentés des fédérations seront étendues au contrôle de la conformité des clôtures et au respect des plans de gestion des enclos. Je voudrais, pour finir, apporter deux précisions juridiques sur la rétroactivité de la loi et sur la création d'une contravention de cinquième classe pour la protection de la propriété privée. La rétroactivité de la loi était nécessaire, car légiférer pour l'avenir aurait fait courir le risque d'une fuite en avant de l'engrillagement, comme on le constate depuis que ce sujet a été médiatisé. Cette rétroactivité doit être aussi importante que possible, pour revenir sur la dégradation des milieux naturels qui est constatée dans plusieurs régions. La proposition de loi porte la volonté de restaurer les corridors biologiques, mais, dans le respect de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, il est nécessaire qu'elle soit limitée dans le temps, proportionnée et justifiée par un motif d'intérêt général suffisant. C'est pourquoi la référence à la loi du 23 février 2005, qui avait accordé un certain nombre de dérogations aux enclos, a été retenue. Par ailleurs, le texte ne remet pas en cause le droit de se clore, mais le conditionne à la libre circulation de la faune et préserve la possibilité d'ériger des barrières plus importantes pour la protection des cultures, des forêts et du domicile, jusqu'à cent cinquante mètres autour de celui-ci, soit un parc d'un peu plus de sept hectares. Par ailleurs, cet abaissement des clôtures est compensé par la création d'une contravention de cinquième classe en cas de violation de la propriété rurale et forestière. Je tiens à préciser qu'il ne s'agit donc pas d'un délit et que le prononcé de cette contravention est dans la main des juges, qui sauront faire preuve de discernement et de sagesse. La commission a donc estimé que la sanction présentait les garanties nécessaires au regard des craintes qui ont pu s'exprimer. Je dois ajouter que, lors des auditions, les associations de terrain en Sologne ont été unanimes pour soutenir cette mesure, car elles constatent des difficultés croissantes liées à la croyance que la nature et ses fruits sont à tout le monde, avant leurs propriétaires et locataires légitimes. Je dois dire que les problèmes posés par ce type de comportement ne s'arrêtent pas, nous le savons bien, aux frontières de cette belle région ! En conclusion, madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, je formule le voeu que le texte qui sera voté ce soir par le Sénat, sous l'impulsion de Jean-Noël Cardoux et de notre commission, permette une réelle avancée, par des mesures efficaces et pragmatiques, et puisse être rapidement repris et largement voté à l'Assemblée nationale. Les amoureux de la Sologne, chasseurs ou non, propriétaires et promeneurs, attendent que cette région retrouve le charme qui a captivé Alain-Fournier, Maurice Genevoix ou Victor Hugo, qui ont porté ses paysages et son atmosphère au niveau de l'art universel. La poésie La poésie a cette force de nous remettre en contact avec le sensible, de nous faire retrouver dans les mots et la rime l'essence de la vie, le goût de la contemplation, de la méditation et de l'imaginaire, un peu comme les amoureux de la nature devant un paysage de Sologne et l'espoir de surprendre un animal. Comme le disait une personne auditionnée, « ici, on aime la chasse, parce que l'on aime la nature ». C'est dans cet esprit que nous avons décidé,

La trame verte et bleue est l'outil qui vise à assurer cette libre circulation. Elle est portée sur les documents d'urbanisme au niveau régional et, plus finement, dans les plans locaux d'urbanisme. En son sein, tout aménagement nouveau devrait être écologiquement transparent. Nous avons beaucoup progressé sur ce point, avec, par exemple, le développement développement des passages à faune, mais il reste nombre de points noirs à résorber. La future stratégie nationale pour la biodiversité, que je vous présenterai dans quelques semaines, traitera largement de ce sujet. Ces efforts ne sauraient être entravés par le phénomène insidieux de l'engrillagement.

pour le faire connaître et le documenter. Le troisième impact porte sur la capacité à lutter contre les incendies, car l'engrillagement peut entraver la circulation des engins de secours. Le risque d'incendie

en ce sens, à certaines des critiques qui visent la chasse en enclos et nous appelle sans doute à aller plus loin, en incitant, notamment, les établissements concernés à adopter des pratiques différentes. L'article L'article 1 de la proposition de loi crée, d'une part, une obligation de mise en conformité des clôtures installées postérieurement à l'année 2005 dans les seules continuités écologiques identifiées dans la trame verte ; il interdit, d'autre part, l'installation de nouvelles clôtures étanches dans l'espace naturel. Je souscris totalement à cette approche, laquelle ne permet toutefois de couvrir que certaines des situations auxquelles nous voulons mettre un terme. Nous ne disposons pas actuellement d'une cartographie des différents types de clôtures avant et après 2005. Il est donc très difficile d'apprécier d'apprécier l'effet de cette mesure et de déterminer si elle sera suffisante. On sait toutefois qu'elle agira sur une partie importante de la Sologne. C'est le premier des objets de cette proposition de loi,

de pénaliser fortement l'intrusion sur le terrain d'autrui. Cette mobilisation de l'écocontribution ne peut s'entendre que dans un projet global de renforcement de la qualité de ces milieux, ce que la rédaction de votre commission a bien pris en compte, et je vous en remercie.

pourront être effectués dans les enclos autour des habitations. Il est évidemment nécessaire de respecter le domicile de chacun, donc de bien les proportionner. Pour autant, cela ne doit pas conduire à soustraire des surfaces entières au contrôle de l'activité de chasse. Il était donc pertinent de disposer de règles claires et différenciées pour deux types

discussion sur ce texte appelle à mon sens plusieurs points de vigilance, concernant, tout d'abord, la prévention des dégâts agricoles et forestiers. En effet, le grand gibier, lorsqu'il est surabondant, cause des dégâts ou ou menace la régénération des forêts, et l'enlèvement de ces grillages ne doit pas accentuer ces problèmes en périphérie des espaces concernés. Nous y serons vigilants. Dans cet esprit, j'estime également que nous devons supprimer, ou restreindre le plus possible, les lâchers de gibier. Je prendrai prochainement des mesures réglementaires, en ce sens : un décret renforcera l'obligation de respecter une densité maximale de sangliers dans les enclos. Ce texte a déjà fait l'objet d'une concertation avec les acteurs ; au-delà d'un animal par hectare, il s'agit d'élevage, et les règles à appliquer doivent donc en tenir compte. Interdire la surdensité est une façon de dissuader l'engrillagement, et cela me semble conforme à une certaine éthique de ces chasses, que nous appelons de nos voeux. voeux. Évidemment, ce décret doit renforcer les mesures sanitaires, avec la mise en place de quarantaines et de plans de gestion des animaux introduits dans les enclos ; dans le cadre des chasses commerciales, un dispositif de marquage des animaux sera également rendu obligatoire.

se trouverait en grande partie dans la volonté de propriétaires privés de créer des enclos de chasse sur leurs parcelles, l'édification de « clôtures imperméables au passage de l'homme et des mammifères

ces enclos « participent à la fragmentation des habitats, notamment forestiers, très présents en Sologne ». Il ajoutait : « L'effet environnemental direct des clôtures, le plus notoire sur l'environnement, s'exerce sur les possibilités de déplacements des grands animaux sauvages, favorisent leur densité, induisent du piétinement, limitent l'apport de nutriments aux sols, accroissent la dégradation du couvert forestier et la prédation directe sur de nombreuses espèces. [ ...] « Les clôtures hermétiques, incluant des grilles à mailles fines en parties basses, affectent également le déplacement et la prise en compte d'autres impératifs biologiques que sont l'alimentation et la reproduction d'autres espèces », notamment la survie des des jeunes bêtes par séparation des parents en raison de clôtures, « mais aussi la circulation de toute la petite faune ». En résumé, « tout concourt à démontrer que les enclos hermétiques ou l'utilisation de grillages imperméables à la faune sauvage sont un non-sens cynégétique, présentent des non-conformités en matière de droit de l'environnement, de droit de l'urbanisme ou de droit rural et échappent partiellement au contrôle des élus et de l'État sur des interprétations juridiques discutables. « Ces pratiques d'accaparement ou de perturbation de l'espace naturel et de l'espace public ne sont plus acceptables.

texte doit donc mettre fin à la prolifération des engrillagements délimitant les propriétés, tout en permettant le maintien des clôtures anciennes réalisées avant la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, qui avait fixé certaines règles. Il doit limiter les enclos au sens strict du terme sans interdire les clôtures végétales ou traditionnelles, assurer la libre circulation des animaux sauvages dans l'espace naturel, notamment sur les trames verte et bleue, assurer le respect des propriétés rurales ou forestières privées par les promeneurs et inciter au désengrillagement en mobilisant l'écocontribution.

L'article 1 précise par exemple que les clôtures, à moins d'être nécessaires à l'activité agricole ou forestière, doivent permettre en tout temps la libre circulation des animaux sauvages. Malheureusement, je le répète, ces nouvelles règles ne s'appliqueront pas aux clôtures datant d'avant la publication de la loi du 23 février 2005. La preuve de l'antériorité de la La preuve de l'antériorité de la clôture pourra être apportée par une attestation administrative. On peut s'interroger sur le rôle des maires. S'ils sont sollicités pour établir une telle antériorité, ils pourront se trouver en difficulté pour en apprécier les preuves. Dans certains cas, ils pourront aussi être de connivence avec le demandeur. Quant au délai de mise en conformité, il a été ramené de dix ans à sept ans. Il ressort de ces différents points que des enclos ne respectant pas ces règles et ayant été édifiés après 2005 pourraient être démontés s'ils n'étaient pas mis en conformité avec la nouvelle législation dans le temps imparti.

de contrôler les enclos antérieurs à 2005 qui subsisteraient, mais qui auront rejoint le droit commun de la chasse, sans se voir opposer l'assimilation de l'espace enclos à un domicile, comme c'est le cas actuellement, ce qui nuit à leur capacité d'action. Concrètement, de telles dispositions interdisent toute intrusion dans ces espaces clos. suivants détaillent les limitations apportées aux lâchers de gibier et les sanctions en cas de non-respect des règles d'agrainage. Ils étendent également le pouvoir des gardes-chasses par la possibilité de dresser procès-verbal en cas de non-conformité des clôtures implantées. L'article 4 crée la possibilité- et non l'obligation -de contribution de l'OFB à la mise en conformité des clôtures existantes non conformes à l'article 1 du présent texte. Cette faculté est étendue aux clôtures antérieures à 2005, ce qui n'était pas le cas initialement, afin d'inciter les propriétaires concernés à ouvrir leurs enclos et à rétablir les continuités.

Sinon, l'engrillagement risque de progresser à une cadence encore plus soutenue, les intéressés partant du principe que tout ce qu'ils auront pu ériger avant l'adoption d'une une nouvelle loi sera de toute façon difficile à détruire.

quelques années, la prise de conscience écologique a transcendé les partis dits « républicains » : de ce fait, la lutte pour la sauvegarde de la biodiversité fait partie des enjeux majeurs de ce gouvernement et de sa majorité. Ainsi, le Congrès mondial de la nature, qui s'est tenu tenu à Marseille en septembre 2021, a su voter une vingtaine de motions pour la sauvegarde de la biodiversité. Rappelons qu'il a réuni près de 20 000 personnes et 1 300 organisations venues de 160 pays.

simplement parce que ce territoire est constitué de forêts propices à la chasse, laquelle prend souvent un caractère privé. De grands propriétaires ont pris l'habitude de clôturer leurs territoires de chasse, ce que le droit français autorise, malgré des effets de bord désastreux pour notre environnement. Cette pratique, face à laquelle nous sommes

Il touche au bien-être animal, porte atteinte à nos paysages et conduit indirectement à de vrais risques sanitaires par la prolifération d'animaux sauvages au sein des enclos. Alors, que faire ? Depuis quelques années, face à la prolifération de ces grillages, les médias,

et comme l'a indiqué en substance Mme la présidente de la commission des affaires économiques, le mieux est l'ennemi du bien. Ce soir, nous ne raviverons pas le débat enflammé et inflammable de la chasse, à quelques semaines d'une échéance électorale de poids : il nous semble que c'est plus sage.

Avant d'entrer plus avant dans le détail de ces dispositions, je souhaite souligner la force de conviction de notre collègue Jean-Noël Cardoux pour faire émerger le sujet. Je tiens aussi à saluer l'important travail réalisé par notre rapporteur, Laurent Somon, afin de trouver les justes équilibres. Le constat

Elle seule peut garantir le brassage indispensable pour éviter la consanguinité et d'autres problèmes sanitaires. Les clôtures ne doivent donc pas être des obstacles.

Il est primordial de garantir la continuité écologique. C'est d'ailleurs toute l'ambition de l'article 1, qui contient une définition claire de la clôture et de ses caractéristiques, tout en adaptant ces dernières aux exigences de la trame verte.

la secrétaire d'État, mes chers collègues, à mon tour, je tiens à remercier notre collègue Jean-Noël Cardoux de son initiative et de l'inscription à l'ordre du jour de notre assemblée de sa proposition de loi visant à modifier les règles d'engrillagement des espaces naturels. seulement à notre conception de l'éthique de la chasse, mais à l'idée de la chasse que nous défendons, ici, au Sénat. Ce problème, particulièrement prégnant en Sologne, au point que l'on en vient à parler de « solognisation », s'étend désormais à d'autres régions de France, où l'on assiste au développement incontrôlé des clôtures. S'il résulte, pour une large part, de la création d'enclos de chasse et s'il protège la propriété privée, il constitue néanmoins un frein à la libre circulation de la faune sauvage. La création des enclos de chasse n'est pas nouvelle : elle est permise par une loi de 1844. Mais le phénomène s'est développé dans les années 1990 et a connu une accélération à partir de 2005.

la non-participation aux remboursements des dégâts de gibier ou encore la faculté de chasser toute l'année quelles que soient les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse. Enfin, depuis que le sujet de l'engrillagement est médiatisé et que des associations se mobilisent, un nouveau mouvement d'accélération a été constaté sur le terrain. Aujourd'hui, la multiplication de ces clôtures, imperméables au passage de l'homme et des animaux, pose de nombreux problèmes.

Comme toujours au sein du groupe Les Républicains, nous sommes résolument tournés vers une écologie, non pas punitive, Aussi, cette proposition de loi prohibe les clôtures ne permettant pas la libre circulation de la faune, c'est-à-dire celles de plus d'un mètre vingt de hauteur, enterrées dans le sol. De plus, elle impose que ces clôtures soient en matériaux naturels ou traditionnels. une norme nationale claire doit être édictée. Cette nouvelle norme s'imposera aux clôtures érigées à compter de la loi de 2005 précédemment citée.

elle le soumet à la libre circulation de la faune. Elle préserve ainsi la possibilité d'ériger des clôtures plus hautes dans certains cas, par exemple jusqu'à cent cinquante mètres autour du domicile.

des clôtures qui seront autorisées. Elles devront permettre d'assurer la circulation de la petite faune. De plus, elles ne devront pas blesser les animaux qui tentent de les franchir ou constituer des pièges pour le gibier.

Je remercie également notre rapporteur, Laurent Somon, qui a mené un travail constructif. Par ses amendements, il a su introduire des évolutions utiles et appropriées visant à mieux encadrer l'engrillagement des forêts françaises.

forêt ne sont plus réservés au sud de la France : ils peuvent se déclarer partout dans notre pays. Or les enclos rendent certaines parcelles inaccessibles aux pompiers. L'interdiction d'ériger des clôtures est donc une mesure salutaire. Elle permettra d'agir sur les continuités écologiques,

cerfs, de chevreuils, de mouflons et de daims. Ces espaces clos quadrillés de miradors, de points d'eau et de points de nourrissage permettent une sorte de safari à l'encontre d'animaux issus d'élevage, souvent importés de Pologne ou de Hongrie. Cela pose des questions d'éthique de la chasse, même les chasseurs en conviennent. Et je ne reviens pas sur l'importation d'espèces exogènes, lesquelles, en s'échappant, peuvent s'hybrider avec des espèces locales et entraîner une pollution génétique. Le second point concerne la pratique dite « de l'agrainage et de l'affouragement », qui n'est malheureusement pas abordée dans ce texte. Cette pratique en enclos ressemble comme deux gouttes d'eau à de l'élevage.

Reconnaissons-le, une telle prolifération est surprenante. Si le nourrissage n'en est pas l'unique raison, il y participe. Aussi, afin de compléter le texte de cette proposition de loi, j'ai déposé deux amendements visant à interdire purement et simplement la pratique des chasses en enclos, ainsi que l'agrainage et l'affouragement. Ce débat ne peut être éludé dans le cadre de nos discussions. Nous attendons également beaucoup des décrets en cours de consultation et de publication. Madame la secrétaire d'État, vous nous avez en partie rassurés, mais nous attendons des dates précises, car l'horloge tourne, vous le savez aussi bien que moi. Le groupe écologiste votera ce texte, car il marque des avancées non négligeables en faveur de la protection de la biodiversité et des paysages. Toutefois, il mériterait d'être complété.

On parle désormais de « solognisation » de tout le territoire. Or cette pratique fait obstacle aux continuités écologiques, pose des problèmes de sécurité incendie et de sécurité sanitaire, empêche la libre circulation de la faune, cantonne les populations de gibier à l'intérieur des domaines, interdit la promenade et nuit au développement du tourisme rural. L'effet environnemental direct des clôtures, c'est-à-dire l'effet le plus notoire sur l'environnement, s'exerce sur les possibilités de déplacements des grands animaux sauvages. L'engrillagement favorise leur densité, induisant du piétinement, limitant l'apport de nutriments aux sols accroissant de fait la dégradation du couvert forestier et la prédation directe de nombreuses espèces. Pis, comme le souligne le rapport de la mission d'information sur l'engrillagement en Sologne, « il s'agit d'une appropriation renforcée de l'espace et un frein à l'exercice de la police de l'environnement, par une déviance du droit des enclos créant des zones de non-droit, où la gestion " cynégétique " est littéralement aberrante Le rapport mentionne même des installations de miradors et postes de tir mettant en danger les usagers des voies publiques. C'est pourquoi l'apparition d'un nouveau type de clôtures, qui ne servait plus à tenir le bétail à l'écart des parcelles cultivées, a suscité une levée de boucliers de la part de nombreux élus, mais aussi des riverains chasseurs et non-chasseurs. En effet, l'engrillagement permet la pratique d'une chasse qui, au fond, n'en est plus une. est plus est, elle est réservée à une élite, ce qui nous rappelle que cette activité n'est pas homogène : elle est en réalité clivée socialement et surtout soumise à une réglementation variable selon les types de chasses et de chasseurs. Pour nous, la chasse en enclos contrevient au principe même d'une chasse populaire, acquis de la République, héritière de la Révolution. L'engrillagement de territoires où les animaux sont, de fait, parqués rompt un équilibre fragile, une certaine équité entre l'homme et la nature et le principe même de la chasse. C'est pourquoi cette proposition de loi est bienvenue. En outre, ces barrières entraînent des risques sanitaires, de surdensité et de maîtrise des populations et interrogent sur l'égalité d'application du droit de la chasse, ainsi que sur la légalité de certaines pratiques. Certes, le texte aurait pu aller plus loin et interdire la chasse dans les enclos hermétiques, à l'exemple de ce qu'a fait la Wallonie, afin de favoriser une chasse durable, qui respecte la fonctionnalité des écosystèmes, la prise en compte des impératifs biologiques des espèces, qu'il s'agisse de reproduction, de nutrition ou de déplacement, et qui tienne compte du fait que la chasse doit que la chasse doit se dérouler en espace naturel. Toutefois, ce texte vise à étendre le droit commun de la chasse à l'ensemble des territoires sur lesquels la chasse est pratiquée et à renforcer l'accès aux enclos cynégétiques à des fins de contrôles. De plus, le texte de la commission prévoit des sanctions en l'absence de mise en conformité de nouvelles clôtures, qui seront punies de trois ans de prison et de 150 000 euros d'amende. Enfin, la commission a précisé le texte pour garantir que ces clôtures ménagent le passage de la faune au sol et ne blessent pas ou ne piègent pas le gibier, tout en permettant la protection des cultures et les régénérations forestières- la liste n'est pas exhaustive. C'est pourquoi nous voterons en faveur de cette proposition de loi. La parole

je tiens tout d'abord à remercier notre collègue Jean-Noël Cardoux pour le dépôt et l'inscription de cette proposition de loi à l'ordre du jour du Sénat. Son contenu et ses objectifs sont importants et attendus dans les territoires concernés, j'y reviendrai.

Je félicite également le rapporteur du texte, Laurent Somon, qui a su s'emparer du sujet, faire évoluer le texte pour le rendre encore plus complet et lui donner une dimension qui, je l'espère, convaincra aussi les députés, qui se sont récemment inquiétés de la même problématique. L'engrillagement des espaces naturels est un phénomène déjà ancien. Il existe depuis plus de cinquante ans dans ma commune, mais il a tendance à s'accentuer et à contaminer, si j'ose dise, une part de plus en plus importante de notre territoire. La Sologne, souvent prise en exemple, est malheureusement caractéristique de ce phénomène, surtout depuis une dizaine d'années, au cours desquelles se sont développées les Comme d'autres ici, je la connais bien, puisque j'y suis né. Depuis près de trente ans, le développement de l'engrillagement y est dénoncé. Déjà, en 1991, le syndicat mixte de la Sologne, dont j'étais vice-président, pointait du doigt le fait que les clôtures « constituaient un problème pour la circulation du grand gibier, enlaidissaient le paysage, nuisaient à l'image de la Sologne et à son développement touristique et détérioraient la qualité cynégétique des populations ». Aujourd'hui, on compte près de 4 000 kilomètres de grillage en Sologne : c'est plus que le nombre de kilomètres de routes départementales dans mon département du Loir-et-Cher En conséquence, les acteurs de terrain, en particulier le Pays de Grande Sologne, ont lancé en 2011 une concertation, laquelle a conduit au rapport d'Yves Froissart. Ce dernier a pu alimenter l'étude menée à la mi-2019 par le Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux et par le Conseil général de l'environnement et du développement durable, en appui au préfet de la région Centre-Val de Loire. Comme Jean-Noël Cardoux, j'ai pu témoigner lors de la réalisation de ces travaux. Les constats dressés, comme les propositions formulées, ont été essentiels pour la prise de conscience générale autour de ce problème. Ils ont aussi permis d'alimenter la proposition de loi qui nous est aujourd'hui soumise. Les mesures énoncées dans ce rapport, ainsi que celles qui sont reprises dans la proposition de loi, balaient l'ensemble des sujets, ce qui était nécessaire. En effet, nous avons besoin d'une réponse complète, claire et de bon niveau, si nous voulons éviter une course à l'engrillagement avant la date de mise en oeuvre des limitations et interdictions contenues dans le texte. Le développement de l'engrillagement est l'un des symboles de l'évolution de la ruralité dans notre pays, mais aussi de l'accroissement d'une forme d'égoïsme dans notre société. Il caractérise non seulement une défense excessive du droit de propriété et un manque de respect des terrains d'autrui, mais aussi une perte de la culture rurale et cynégétique, ainsi qu'une atteinte à la biodiversité. Notre rapporteur souligne également une forme de dislocation des relations sociales traditionnelles dans les campagnes. L'engrillagement est donc l'une des expressions de cette perte du vivre-ensemble. Malheureusement, il a d'autres conséquences plus palpables et contre lesquelles il faut lutter. Les constats réalisés par la mission de Michel Reffay et de Dominique Stevens sont clairs une fermeture de l'espace qui dégrade la qualité paysagère, la valeur patrimoniale et la fonctionnalité de toute la Sologne et nuit à son image et à sa perception par la société une appropriation renforcée de l'espace et un frein à l'exercice de la police de l'environnement, par une déviance du droit des enclos créant des zones de non-droit où la gestion « cynégétique » est aberrante un risque sanitaire lié à l'introduction d'animaux, au cloisonnement des populations, à la fragmentation des habitats, à la surpopulation manifeste de certains enclos et parcs, sans contrôle vétérinaire une entrave à la libre circulation des grands animaux sauvages, avec des conséquences sur les populations animales, les types de chasse pratiqués et, indirectement, les habitats naturels des problèmes de sécurité routière induits par la canalisation des grands animaux du fait des clôtures, avec une suraccidentalité ; des dégâts dus au gibier concentré sur les propriétés non closes une mise en péril de l'état forestier en présence de surpopulation de suidés et cervidés ; enfin, des installations de miradors et postes de tir mettant en danger les usagers des voies publiques. La proposition de loi visant à limiter l'engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée que nous examinons tend à poser des règles pour mettre fin à ces difficultés, avec pour conséquence l'amélioration de la sécurité incendie, la protection de la sécurité sanitaire, l'arrêt de la destruction de la faune et de la flore, ainsi que le développement du tourisme rural. Les différentes mesures proposées sont globales et vont dans la bonne direction : l'interdiction des clôtures ne laissant pas passer la faune et n'utilisant pas des matériaux naturels est au coeur de ce texte. Il s'agit finalement de redonner de l'air à nos campagnes et à nos forêts, sans priver les propriétaires de leur bien. Je proposerai d'ailleurs, par voie d'amendement, d'aller encore un peu plus loin en interdisant les merlons de terre longeant nos routes.

ont les mêmes conséquences néfastes pour la faune, pour le patrimoine naturel et pour le paysage que les clôtures que nous interdisons. L'abaissement des clôtures postérieures à 2005 permet de contourner le phénomène d'opportunité, que l'on a pu constater, visant à engrillager rapidement, par peur de la nouvelle réglementation. Les exceptions prévues et recalibrées par le rapporteur étaient aussi importantes. Les mesures d'accompagnement que sont l'utilisation de l'écocontribution pour financer les continuités écologiques, le délai de mise en conformité de sept ans et la contravention de violation de propriété permettent d'équilibrer le texte et les mesures d'interdiction précédentes. Ces compensations doivent créer les conditions d'acceptabilité de ce texte pour les propriétaires. Enfin, les apports de la commission des affaires économiques concernant les contrôles de l'intérieur des enclos par les agents de l'OFB, l'Office français de la biodiversité, et des clôtures par les agents assermentés des fédérations me semblent également aller dans le bon sens.

après avoir rappelé que la gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats relève de l'intérêt général, l'article L. 420-1 du code de l'environnement prévoit que « les chasseurs contribuent au maintien, à la restauration et à la gestion équilibrée des écosystèmes en vue de la préservation de la biodiversité Or une pratique de la chasse contraire à ces principes se répand et s'aggrave ces dernières années : des milliers de kilomètres de clôtures sont érigés dans les milieux naturels, empêchant la libre circulation des animaux sauvages et méconnaissant les dispositions relatives à la continuité écologique. En Sologne, le territoire se trouve morcelé, en pleine zone Natura 2000, la plus importante par sa taille au niveau européen, et l'attractivité du territoire s'en voit affectée. Dans certains domaines privés de chasse, on trouve des animaux provenant d'élevages à forte concentration. Il n'y a donc plus, pour le chasseur, de recherche du gibier, plus d'acte de chasse à proprement parler. Le président de la Fédération nationale des chasseurs a même évoqué le massacre de 300 sangliers et cervidés en trois heures dans un enclos. Je suis chasseur, mais je ne me retrouve pas dans ces pratiques.

qui s'applique dans les enclos cynégétiques, permettant de chasser le gibier à poil sans limitation du nombre de prélèvements et à tous moments. S'il est légitime d'ériger des clôtures autour d'une habitation pour protéger la propriété privée, l'extension du « privilège de l'enclos » sur des terrains de plus en plus vastes, qui bénéficie aux chasses commerciales, est inacceptable. Il s'agit d'une forme de confiscation des animaux sauvages, lesquels, par essence, n'appartiennent à personne. Le législateur ne peut pas fermer les yeux sur ce massacre de la faune et du paysage.

le Centre-Val de Loire a tenté, en 2018, de faire cesser ce développement anarchique, en encadrant la hauteur et les caractéristiques des clôtures. cela peut contribuer à freiner l'apparition de nouvelles clôtures, celles qui existent et le « privilège de l'enclos » ne peuvent être remises en cause sans une modification de la loi. Certains proposent d'aller plus loin et d'interdire toute chasse en enclos. Pourquoi pas ?

avec une rétroactivité de la loi limitée et proportionnée. L'article 4 du texte permet d'accompagner financièrement le remplacement des clôtures par des haies. Les enclos antérieurs au 23 février 2005 auraient pu être concernés par la mise en conformité à des normes les rendant compatibles avec la protection de l'environnement et des paysages. Néanmoins, dans un premier temps, la démarche de l'auteur de la proposition de loi me semble aller dans le sens d'une meilleure sécurité juridique. À ce stade,

concurrentes à l'Assemblée nationale, et j'invite nos collègues députés à se saisir de ce texte sans attendre, afin que ces mesures puissent s'appliquer au plus vite. En effet, un délai de sept ans est d'ores et déjà prévu pour la mise en conformité.

faire face au développement inquiétant des clôtures grillagées en forêt, tout en protégeant mieux la propriété privée. Trop souvent, cet engrillagement résulte de la création d'enclos de chasse, qui constituent un frein à la circulation de la faune sauvage. C'est assez simple à comprendre : si vous empêchez le gibier de sortir d'un espace, vous l'empêchez également d'y entrer, donc de s'y alimenter et de s'y reproduire. Nous connaissions la problématique de l'artificialisation des sols, nous devons désormais prendre note du développement croissant de cet engrillagement. On pourrait me rétorquer que ces enclos sont rarement efficaces à 100 % et qu'ils ont très souvent des failles qui permettent, du moins à certaines espèces, de circuler. Or une telle situation est tout aussi inquiétante !

Notons par ailleurs que ces parcs de chasse à caractère commercial ne participent pas aux remboursements des dégâts causés aux agriculteurs. Le développement de cette activité, au détriment des fédérations de chasse, pourrait nuire à ce budget si important pour nos cultivateurs, mais aussi pour les chasseurs attachés à préserver le sens même de leur passion, à savoir la régulation. Notons aussi que ces parcs bénéficient aujourd'hui d'une exemption de plan de chasse. En effet, ils peuvent ne pas respecter les dates d'ouverture et de fermeture, ce qui ne correspond pas à l'idée que je me fais de cette pratique, qui doit rester populaire et connectée à son environnement. Vous l'aurez compris, je salue ici la volonté du texte de supprimer ces dérogations, afin de garantir une chasse responsable. Enfin, il arrive cependant que cet engrillagement soit une réponse au non-respect de la propriété privée. En effet, certains néoruraux oublient qu'un espace forestier peut être une propriété privée et qu'il n'existe pas un droit à s'y promener en dehors des chemins ruraux. observait autrefois une large tolérance. Hélas, de plus en plus de tensions naissent. Le développement de certaines pratiques, comme le quad ou le passage répété de vététistes, nuit aux différentes espèces et aux plantations, dégradant la propriété elle-même. Cette proposition de loi entend rappeler que le droit de propriété a valeur constitutionnelle. Elle crée ainsi une amende de 1 500 euros pour le fait de pénétrer sans autorisation dans une propriété rurale ou forestière. Il est important de le rappeler, mes chers collègues, car ces clôtures, lorsqu'elles sont installées par des particuliers, le sont non pas par plaisir, mais par nécessité. Elles ont un coût important, dénaturent souvent les paysages et, surtout, peuvent freiner l'avancée des pompiers en cas de feu de forêt. Je pense ici bien sûr à mon département du Gard, mais aussi aux autres départements du sud de la France. De fait, je crois utile de le préciser, pour ce qui concerne les clôtures existantes, les propriétaires auront sept ans pour se mettre en conformité avec les dispositions du texte. clôtures d'intérêt public, par exemple autour des chemins de fer et des aéroports, ou encore les clôtures agricoles, resteront autorisées. Précisons également que l'écocontribution pourra être utilisée pour effacer les clôtures et les remplacer par des haies. Cette proposition de loi est donc un juste équilibre entre préservation de la continuité écologique et respect du droit de propriété, lequel est parfois méconnu, avec une confusion entre droit à proprement parler et tolérance. Au travers de ce texte, nous faisons toute la lumière sur cette notion, ce qui ne semble pas inutile, afin d'apaiser certaines relations dans le monde rural. Je tiens à saluer ici le travail de notre collègue rapporteur, Laurent Somon, qui a su préserver un consensus, tout en apportant des précisions utiles, afin de nous assurer la bonne application du texte. Enfin, je veux remercier chaleureusement notre collègue Jean-Noël Cardoux d'avoir pris à bras-le-corps cette problématique et d'avoir su conjuguer mesure, sens de l'écoute et détermination.

Cet amendement est conforme à notre politique en faveur de la préservation de la biodiversité visant à maintenir et à remettre en bon état les continuités écologiques. Quel est l'avis de la

Ceux-ci, par exemple autour des demeures historiques, sont devenus des attractions touristiques attirant un grand nombre de visiteurs et nécessitant des investissements importants. Si certains jardins sont déjà clos de murs, d'autres sont directement ouverts sur des forêts. Il s'agit donc de les préserver des dégâts de gibier, mais aussi de participer à l'essor économique de ces sites et à la valorisation du patrimoine.

sangliers et cervidés contenus dans les espaces clos à visée cynégétique sont souvent responsables de dégâts dans notre biodiversité et sur nos espaces agricoles. Par cet amendement, nous demandons donc aux propriétaires de procéder à la mise en conformité de leurs clôtures en veillant spécifiquement à la protection des équilibres écologiques et des activités agricoles ou forestières du territoire

Or j'aimerais épargner aux maires des pressions supplémentaires. Nous estimons que le propriétaire doit apporter par lui-même des preuves d'antériorité en s'appuyant en priorité sur des documents d'urbanisme qu'il a en sa possession ou qu'il obtient à l'issue d'une recherche. Je voudrais à tout le moins avoir la certitude que l'attestation administrative,

justement fait observer M. le rapporteur, il existe une preuve très simple que les directions départementales des territoires ou les fédérations départementales des chasseurs pourront apporter. En effet,

comprenant les infrastructures, le matériel de production, d'élevage ou de transformation ou les entrepôts de livraison inhérents à l'activité agricole ou forestière. L'ajout de la notion de siège d'exploitation est une précaution indispensable pour répondre aux exigences de sécurité en milieu naturel des personnes, des animaux et des biens.

Bernard Buis. Les zones de non-droit ne sont pas forcément celles que l'on croit. Le manque de contrôle au sein de ces enclos fermés est particulièrement problématique. Il se révèle donc indispensable de renforcer les pouvoirs de la police de l'environnement. En complément de l'article 1 adopté en commission, nous proposons de faciliter les contrôles mis en place par les fonctionnaires et agents chargés de cette mission, en leur permettant d'effectuer leurs inspections à tout moment. Quel est l'avis de la commission ? L'amendement

Par ailleurs, comme vous le savez, après consultation des administrations concernées, la commission a bien traité ce point en introduisant dans le texte l'article 1 , qui donne pouvoir à l'OFB de contrôler les enclos clos-

Quelques rares exceptions pourraient être justifiées, mais les exceptions amènent trop souvent leur lot de dérives. Voilà pourquoi je propose une interdiction claire et nette, qui fera émerger, je n'en doute pas, d'autres solutions pour les quelques cas où l'agrainage et l'affouragement pourraient avoir un intérêt.

paraît assez irréaliste et peu pragmatique au regard des besoins de protection des cultures et de l'importance des dégâts de grand gibier ici ou là, comme vous l'avez dit. L'article L. 425-5 du code de l'environnement interdit déjà le nourrissage en vue de concentrer territoire et n'autorise que les opérations d'agrainage dissuasives en fonction des besoins locaux et dans le respect du schéma départemental de gestion cynégétique, auquel seront désormais soumis les différents enclos.

j'avais pris l'initiative, en accord avec Mme Wargon, de présenter un amendement, adopté par le Sénat, visant à interdire le nourrissage en tas en vue d'attirer le gibier,

: La parole est à M. le rapporteur. La proposition de loi modifiée par la commission prévoit que les agents de développement assermentés des fédérations de chasseurs pourront désormais constater par procès-verbaux les infractions relatives à la conformité des clôtures implantées dans les espaces naturels,

de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique (texte de